La séance est reprise. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois nécessaire, alors que le processus d'élaboration des lois suscite de nombreuses questions, de rappeler solennellement quelques-uns des principes de notre République. La Constitution du 4 octobre 1958 dispose, à l'article 24, que « le Parlement vote la loi

est examiné successivement dans les deux Assemblées [ ...] en vue de l'adoption d'un texte identique ». Le pouvoir législatif appartient donc au Parlement et à lui seul. Aucune

Aucune commission, aucun comité d'experts dépourvu de légitimité démocratique n'est habilité à réécrire un texte de loi en cours de navette. C'est le rôle du seul Parlement d'amender les textes de loi qui lui sont soumis, par l'exercice du droit d'amendement, lequel appartient à chacun d'entre vous, comme parlementaire. Le Parlement est composé de deux assemblées qui détiennent exactement les mêmes prérogatives dans l'initiative et l'élaboration de la loi, l'Assemblée nationale ne pouvant statuer définitivement qu'après échec éventuel de la commission mixte paritaire et une nouvelle lecture dans chaque assemblée. Je dois donc rappeler aux groupes de la majorité de l'Assemblée nationale que la proposition de loi dont ils souhaitent travailler à la réécriture partielle a été transmise au Sénat depuis le mardi 24 novembre dernier, après que les députés l'ont adoptée. Il revient donc au Sénat, et à lui seul, de l'examiner et de réécrire, si cela se révélait nécessaire, une ou plusieurs de ses dispositions. Après l'examen du texte par le Sénat, il reviendra alors au Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire ou de décider la poursuite de la navette parlementaire en prévoyant une deuxième lecture

La situation démontre une fois de plus qu'avoir deux chambres est un atout, dans une démocratie. Bien sûr ! C'est d'autant plus heureux qu'il existe au Sénat une longue tradition d'équilibre entre la protection de nos concitoyens et le respect des libertés publiques. L'urgence est donc de revenir, dans les mots et dans les faits, à un fonctionnement normal de nos institutions et de respecter, tout simplement, les procédures constitutionnelles. Voilà ce que je voulais dire solennellement en ce début de séance.

Monsieur le ministre, la « ferme France » va mal, je ne vous apprends rien. On constate une baisse générale de la production et des volumes, une baisse significative de la valeur ainsi qu'une baisse des effectifs, tant chez les exploitants que chez les salariés. Sans les aides de la politique agricole commune (PAC) et de l'État, un agriculteur sur deux n'aurait pas de revenus.

; enfin, la folie des surtranspositions- j'y insiste ! -, qui vise à supprimer des techniques ou à imposer des normes toujours plus contraignantes, sans calcul d'impact sur les revenus de nos exploitants comme de nos transformateurs.

Imposer toujours plus de contraintes à notre agriculture conventionnelle sans augmenter les prix de vente, en raison de la pression des cours mondiaux ou de contrats de type Mercosur, condamnera nos agriculteurs. Les consommateurs sont-ils pour autant prêts à payer plus cher et à perdre du pouvoir d'achat ? Je n'en suis pas L'agriculture conventionnelle a donc toute sa place et je reste persuadé qu'elle est beaucoup plus qualitative que celle que l'on importe et que l'on ne contrôle pas. Monsieur le ministre, j'attends que vous apportiez des réponses précises à ces questions Revenons au budget, qui est, je le rappelle, financé par l'Union européenne et par la France. Alors que vous êtes en pleine négociation sur la PAC, vous nous avez indiqué vouloir suivre la période passée, mais je vous rappelle que nous avons supporté des corrections européennes considérables, nous avons fait subir aux agriculteurs des retards de paiement de leurs subventions, nous avons été obligés de transférer des fonds vers le Fonds européen agricole pour le Nous n'avons pas traité le problème de l'installation. Nous demeurons sans réponse structurée à la question très grave des aléas de toutes sortes qui insécurisent nos agriculteurs. Pendant ce temps, nous avons élevé nos exigences environnementales sans nous en donner les moyens. Tout cela se trouve au coeur de notre discussion budgétaire et nous aurons l'occasion d'y revenir. Les agriculteurs sont satisfaits du retour à des paiements à meilleure date, nous vous donnons acte. Toutefois, je dois confesser n'être pas tout à fait sûr que les conditions dans lesquelles ont été engagés des crédits au cours de la période allant de juin 2019 à juin 2020, avec des engagements massifs, nous garantissent contre de futures déconvenues. Nous avons parlé des corrections financières européennes, j'ai aussi en tête les désengagements considérables d'autorisations d'engagement intervenues ces dernières années. Pour le reste,

avez tenus lors de la récente réunion avec les parlementaires sur la politique agricole commune rejoignent largement le diagnostic que nous établissons sur le défaut de cohérence entre les objectifs agricoles et les outils prévus pour les atteindre. atteindre. Je confesse là encore en avoir été surpris, même inquiet, non seulement parce qu'ils étaient presque un aveu d'échec, mais surtout parce qu'ils en ont annoncé le renouvellement à l'avenir. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué être satisfait de la nouvelle PAC, dans son aspect tant budgétaire que réglementaire. Le succès budgétaire est tout de même très relatif, puisque, hors plan de relance européen, les dotations du Feader sont vouées à baisser. C'est très préoccupant au regard d'un objectif combiné de souveraineté alimentaire et de transition agroécologique. Certaines Certaines estimations font état d'une perte de production liée à la future PAC pouvant atteindre des niveaux très significatifs. Moins de production en perspective et moins d'aides : l'équation sera très difficile à résoudre

ministre, vous m'avez surtout surpris quand vous avez évoqué la création de valeur comme issue indépassable d'une politique agricole soutenable. En même temps, vous avez condamné l'attitude consistant à exiger des agriculteurs une réorientation de 30 % de leur production du fait de la transition agroécologique.

la future PAC des ? Vous avez affirmé que le budget ne devait pas contraindre la politique et que l'instrument ne devait pas prévaloir sur l'objectif. Nous pouvons partager ce point de vue. C'est la raison pour laquelle, ayant estimé que votre projet de budget ne servait pas des objectifs qu'il vous faudra préciser,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos productions agricole et forestière, ainsi que nos entreprises de pêche ne se sortent pas d'une crise, plus ou moins larvée, qui dure depuis des années et que l'année en cours portera sans doute à son comble. En effet, la plupart des secteurs sont touchés. en tant qu'élu d'un territoire d'élevage, ne pas témoigner, à titre d'illustration, des situations dramatiques de l'élevage bovin allaitant, qui nécessitent des interventions urgentes, mais aussi des accompagnements de plus long terme, pour donner des perspectives aux exploitants ? Les différentes lois de finances, initiale et rectificatives, applicables en 2020 n'ont pas apporté de réponses convaincantes à cette situation et le projet de budget pour 2021 dédié à la mission

Le plan de relance derrière lequel le Gouvernement tend à s'abriter est une opération à un coup qui prétend pourtant porter une modification durable de nos capacités agricoles orientée vers la souveraineté alimentaire et une agriculture plus écologique. Il ne s'appuie sur aucune évaluation de son efficacité au long cours. D'un point de vue budgétaire, des engagements conjoncturels ne peuvent fonder une transformation de l'agriculture vers des modes de production structurellement différents répondant aux enjeux écologiques et sociaux, tout en assurant un modèle économique viable qui garantisse aux agriculteurs un revenu décent. Cela demande du temps et des soutiens opiniâtres. Monsieur le ministre, vous avez évoqué une agriculture créatrice de valeur et, en même temps, moins dépendante du marché. Vous êtes allé jusqu'à regretter que certains veuillent imposer des contraintes environnementales aux exploitants et vous vous réjouissez d'avoir imposé 20 % au moins de contenu environnemental au premier pilier de la PAC. Reconnaissez-le : il est difficile de vous suivre Nous avons besoin d'objectifs clairs nécessitant de faire des choix clairs et lisibles, donnant le cap à tous les agriculteurs et à toutes les agricultures, permettant aux exploitants de se lancer dans les adaptations nécessaires de leurs systèmes de production.

Ne métropolisez pas l'agriculture française, monsieur le ministre ! Le volet forestier de la mission illustre un manque de visibilité des politiques auxquelles concourent nombre de crédits de la mission. représentent à peine 15 % des concours publics de votre budget et passent de plus en plus par des dépenses fiscales très inégalement profitables pour les forestiers.

Pour en revenir à la forêt, alors que l'actuel contrat d'objectifs et de performance de l'ONF, l'Office national des forêts, arrive à peine à son terme, vous avez décidé de réduire le plafond d'emplois de l'établissement. Contre votre avis, l'Assemblée nationale en a décidé autrement. L'attitude du Gouvernement me paraît peu cohérente avec la volonté affichée d'agir pour la forêt. On ne peut que regretter le décalage permanent entre les discours et les actes, que l'on retrouve également dans votre politique agricole. Je sais bien que l'ONF rencontre des problèmes. Son résultat économique, sensible à l'évolution du prix du bois, qu'il ne maîtrise pas, n'est pas bon et son endettement ne cesse de croître, mais le Gouvernement préfère souvent cette issue à une prise en charge responsable des déséquilibres financiers courants. Monsieur le ministre, l'ONF subit des handicaps sérieux. Il doit supporter un taux de contribution employeur au titre des retraites de ses salariés, sans les aménagements qui profitent à d'autres organismes à vocation industrielle et commerciale, comme Orange.

Le programme 206, « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », connaît une progression de ses crédits. Elle répond essentiellement à des évolutions subies par les conséquences du Brexit, auxquelles le Gouvernement a souhaité répondre en créant des emplois souvent non pourvus, qui soulignent, par contraste, la faiblesse des moyens de contrôle des importations hors Union européenne. De même, nous le voyons bien, les crédits dédiés aux indemnisations des sinistres sanitaires

Pour le reste, les réflexions et réorganisations de notre appareil de maîtrise des risques sanitaires semblent abandonnées, tandis que des points noirs subsistent : déserts vétérinaires en formation, abattoirs publics à l'agonie, restructurations de laboratoires difficiles.

Le Gouvernement a beaucoup communiqué sur la réduction des autorisations de mises sur le marché de produits comprenant du glyphosate. Reste que l'indicateur que vous invoquez ne dit rien du nombre de doses employées. Sur ce sujet, une grande confusion règne. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement effet dû enregistrer la défection de l'Institut Pasteur, pourtant choisi comme lauréat de l'appel à projets pour approfondir les études de toxicité. De votre côté, monsieur le ministre, vous avez déclaré être hésitant sur les suites à donner à l'engagement de campagne d'une sortie du glyphosate. en soit, l'objectif demeure à l'horizon 2023 dans votre projet de budget, mais les moyens n'y sont pas. Ils y sont d'autant moins que vous déshabillez le Casdar de 10 millions d'euros, alors que le solde du compte vous permettrait de l'abonder plus significativement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à voir ce budget sans grande nouveauté, un rapporteur sérieux pourrait penser que tout va bien va bien ! C'est d'autant plus vrai que ce budget comporte plusieurs points satisfaisants, conformes à ce que le Sénat défend depuis longtemps, un maintien du dispositif TO-DE pour deux années supplémentaires - nous l'avions sauvé voilà deux ans et nous nous battons pour sa pérennisation -, une stabilisation du budget des chambres d'agriculture, que nous avons arrachée l'année dernière, vous permettant, monsieur le ministre, de mieux déployer votre politique aujourd'hui, et, surtout, la mise en place d'un volet agricole de 1,2 milliard d'euros dans le plan de relance, pour couvrir des dépenses d'investissement essentielles, que nous avons défendu au sein de la cellule de crise covid du Sénat. Nous nous réjouissons que vous souteniez enfin les aides aux investissements favorables à la réduction d'intrants, au bien-être animal et à la réduction des risques liés aux aléas climatiques. Depuis deux ans, le Sénat réclamait ces mesures, tandis que le Gouvernement s'y opposait. Toutefois, ce budget comporte trois vices, qui sautent aux yeux et ont failli nous aveugler, un peu comme la lettre volée a failli aveugler le détective Auguste Dupin d'Edgar Allan Poe. Le premier vice concerne les aides de crise liées au confinement. Elles ont été promises au mois de mai dernier. Pourtant, aucune aide nationale n'a été versée à ce stade. Seules les aides européennes pour la distillation de crise de la viticulture ont été versées. Depuis le début de la crise au mois de mars dernier, les producteurs n'ont encore rien reçu. Est-ce ainsi que vous pensez répondre à l'urgence ?

Le deuxième vice concerne la sincérité du budget. Par exemple, vous promettez 7 millions d'euros pour la recherche sur le glyphosate et 7 millions d'euros pour la recherche sur les betteraves. Où sont-ils dans ce budget ?

Par un tour de passe-passe budgétaire, vous vous apprêtez à spolier les cotisations des agriculteurs destinées à financer une recherche qui leur revient. Vous prônez la recherche de solutions à tout-va pour accélérer les transitions et, dans

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je rejoins l'analyse de Laurent Duplomb et souhaite, en complément, vous faire part d'autres facteurs d'inquiétude liés au changement climatique et à la sécurité sanitaire. Ce sont des facteurs de risque que le budget que vous proposez ne prend pas suffisamment en compte, monsieur le ministre, ce qu'il faut regretter. Nous constatons, chaque année, sur l'ensemble du territoire français que la nature et la fréquence des aléas climatiques et sanitaires augmentent. J'en veux pour preuve les sécheresses à répétition connues depuis 2016 ou, plus spécifiquement cette année, les impacts très forts sur les rendements de l'épidémie de jaunisse sur les betteraves. Pourtant, chaque année, nous constatons que la provision pour aléa est sous-dotée. Cette année, par exemple, l'État avait prévu une provision de 175 millions d'euros. Il en dépensera finalement 230 millions d'euros, pour compenser les effets de la sécheresse de 2019 et payer les apurements communautaires. Compte tenu des événements que nous avons connus cette année, il est certain que les 15 millions d'euros supplémentaires prévus dans le budget ne suffiront pas à financer les indemnisations liées à la sécheresse de cet été

Je pense à l'influenza aviaire, trois cas ayant été découverts la semaine dernière en France, ou à la tuberculose bovine, dont le nombre de foyers a considérablement augmenté ces dernières années. Je pense également aux risques liés à la peste porcine africaine ou à l'exposition des élevages de visons à la covid-l9. Quelles actions comptez-vous mener sur tous ces points ? Il faut agir vite et fort en matière de prévention, de sensibilisation, de biosécurité. À défaut d'actions vigoureuses, les filières sont exposées au risque que la France perde son statut indemne, ce qui bloquerait les exportations vers de nombreux pays. Tous ces dangers épidémiques font peser des risques forts sur le budget. Pour mémoire, le coût budgétaire de l'épisode H5N8 de 2017 a été estimé à plus de 64 millions d'euros pour le seul programme 206. Selon moi, ces risques ne sont pas suffisamment pris en compte dans le budget présenté.

Monsieur le ministre, à la découverte de ce budget, j'ai d'abord cru à une provocation. Je vous revois à la même place, voilà quelques semaines, lors de l'examen du texte sur les néonicotinoïdes, vanter les mérites de la recherche agricole, seule solution à vos yeux pour trouver des alternatives rapides à ces pesticides.

devons reconnaître que ce grand écart idéologique ne doit pas être confortable pour vous. Sachez qu'il est très problématique pour nos campagnes. Les dépenses du Casdar permettent d'affecter les cotisations des agriculteurs au financement de la recherche agricole appliquée. C'est un système particulièrement vertueux, auquel nous sommes très attachés. Aucun argument technique n'est recevable : la réduction du plafond, même en cas de baisse de l'activité agricole, n'est pas inéluctable. Entre 2014 et 2017, le ministère de l'agriculture maintenait un plafond très au-dessus du niveau des recettes.

Erreur stratégique, car de nombreux projets ne pourront pas être financés. Les instituts techniques nous ont transmis une liste de 47 projets majeurs, refusés ces dernières années, malgré leur intérêt. Erreur stratégique, car les fonds du plan de relance affectés à la recherche sont des fusils à un coup, je vous l'ai déjà dit, monsieur le ministre, alors que la recherche nécessite un temps long et que le défi de la réduction des pesticides ne sera pas relevé en un an.

je vous remercie

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, parce que l'agriculture a démontré une certaine résilience en garantissant le bon déroulement de la chaîne alimentaire durant le premier confinement, nous pourrions avoir le sentiment qu'elle a moins souffert des conséquences de la crise sanitaire.

on peut regretter un budget peu dynamique, alors que l'agriculture doit amplifier sa transition écologique, en plus d'éponger les conséquences de la crise sanitaire. Sans le plan de relance, le Fonds Avenir Bio est simplement reconduit pour 2021, alors que l'on observe un léger décrochage dans le cadre de l'objectif de 15 % de surfaces agricoles cultivées selon un mode biologique d'ici à 2022. Par ailleurs, les crédits relatifs à la pêche sont stables, alors que le Brexit risque de peser sur l'activité des pêcheurs français. Les crédits de la mission « Plan de relance », à hauteur de 390 millions d'euros en crédits de paiement, viennent en renfort, mais sans que l'on sache comment ces moyens, sous tutelle du ministère des comptes publics, s'articuleront avec ceux du ministère de l'agriculture.

afin d'augmenter le plafond de dépenses du compte d'un peu plus de 12 millions d'euros. Le Casdar doit avoir les moyens de sa politique, définie par le Programme national pour le développement agricole et rural.

Il met en particulier l'accent sur les thèmes du développement des circuits courts ou encore la gestion intégrée de la santé animale et végétale. Ces thèmes répondent à des attentes sociétales fortes. Aussi la baisse des crédits du Casdar est-elle un mauvais signal pour ceux qui ont la charge d'encourager la diffusion des systèmes de production innovants, à savoir les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Je salue en revanche l'effort financier réalisé en direction des projets alimentaires territoriaux (PAT), avec une dotation de 80 millions d'euros sur deux ans. Depuis leur création en 2014, les PAT peinent à se multiplier. Alors qu'un objectif de 500 PAT a été fixé pour 2020, nous avons atteint moins de la moitié

Il faut donc les encourager, d'autant qu'ils sont consensuels. Si leur décollage est lent, sans doute convient-il de s'interroger sur leur technicité et flécher une partie des moyens sur leur promotion. Cela implique une simplification et une prise de conscience des élus locaux, sans lesquels rien ne pourra se faire. J'en viens à la gestion des risques agricoles. La réserve pour aléas, portée à 190 millions d'euros pour 2021, risque, une nouvelle fois, de ne pas être à la hauteur des besoins. Cet été, pour répondre aux périodes de sécheresse qui se sont multipliées ainsi qu'aux charges liées aux apurements communautaires, le Fonds national de gestion des risques en agriculture s'est retrouvé sous-doté d'au moins 50 millions d'euros. Avec une augmentation de seulement 15 millions d'euros, on s'oriente vers le même problème, au regard d'aléas climatiques répétitifs.

Il y a urgence à soutenir une quarantaine d'établissements en difficulté, qu'une augmentation de 0,5 % des moyens dans le projet de loi de finances pour 2021 ne suffira pas à sortir

Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes qui se battent au quotidien, simplement pour gagner leur vie et nous nourrir. Nos paysans souffrent. Certains préfèrent mettre fin à leur vie, car les obstacles sont trop grands. On déplore plus de deux suicides par jour, nous ne pouvons pas les oublier. La

Pourtant, certains secteurs ont été durement atteints par cette crise sanitaire, notamment du fait des fermetures dans le secteur de la restauration et des petits commerces. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'agriculture, L'agriculture, qui satisfait pourtant un besoin essentiel, ne représente que 1 % du plan de relance. Alors que le capital et les actionnaires profiteront allègrement de ce plan, les « premiers de corvée », dont les agriculteurs font partie, sont les grands oubliés. Nous le regrettons pensez-vous sincèrement que la baisse de 23 millions d'euros des crédits dédiés à la modernisation et au renouvellement des exploitations est aujourd'hui justifiable ? Que dire aussi de la baisse de 12 millions d'euros du budget consacré à la gestion équilibrée des territoires ? C'est incompréhensible ! De nombreux opérateurs, pourtant essentiels, et du travail (Anses) et l'Agence Bio voient leurs subventions diminuer de 4 millions d'euros, au nom de la « maîtrise des dépenses publiques » ! Monsieur le ministre, nos fonctionnaires- vos équipes ! -ont besoin de moyens humains et financiers pour répondre aux défis qui nous sont posés. Ce budget représente également l'échec des politiques publiques menées jusqu'à présent en matière de transition agroécologique. Cette année, contrairement aux engagements présidentiels, nous ne sommes pas sortis du glyphosate. Pire, vous avez de nouveau autorisé les néonicotinoïdes pour la filière betterave. Le pire, c'est que vous amputez l'enveloppe allouée au Casdar de 10 millions d'euros par rapport à 2020, alors même qu'il s'agit d'un levier pour accompagner la transition agroécologique de notre agriculture. Comment construire des alternatives viables et pérennes, si nous ne donnons pas les moyens à la recherche de les trouver ? Monsieur le ministre, la transition agroécologique est un enjeu essentiel si nous voulons continuer à nourrir l'humanité, tout en préservant notre planète déjà très durement atteinte. C'est un enjeu environnemental, mais également sanitaire et social. Surtout, c'est un enjeu pour nos agricultrices et agriculteurs, pour leur santé, pour la santé des terres qu'elles et ils cultivent, sans qu'ils se retrouvent pour autant dans la misère. Les investissements et les accompagnements sont donc essentiels.

ailleurs, monsieur le ministre, on ne vous entend pas sur un sujet majeur : que pensez-vous des traités de libre-échange ? Il y en a quinze sur la table et on ne connaît pas votre avis ! C'est pourquoi économique et commercial global, ici, au Sénat ? Il est impensable qu'un traité de libre-échange d'une telle ampleur, qui fait courir tant de risques à notre agriculture, mais aussi à nos normes environnementales et sociales et à nos services publics, ne soit toujours pas soumis à la ratification du Parlement dans son ensemble ! Cela est révélateur d'un véritable mépris du Parlement et du processus démocratique de la part du Gouvernement.

mais le risque est que ces aides soient élevées pour les deux prochaines années, et moindres les années suivantes, alors que la crise sociale ne sera pas finie.

Ancienne maire de la commune rurale de Hertzing et actuelle conseillère départementale du canton de Sarrebourg, dans le département de la Moselle, la ruralité me parle : j'y suis née. je rencontre des agriculteurs responsables et imaginatifs. Ils ne comptent pas leurs heures et connaissent tous les risques inhérents à leur métier, qu'il s'agisse de l'état sanitaire de leurs animaux, des attaques parasitaires subies par la forêt ou des rendements catastrophiques par manque d'eau des cultures. sont malgré tout résilients, comme toujours, telles des vigies de notre bien-être et de notre sécurité alimentaire. Durant cette pandémie, ils se sont tus, par décence, souhaitant privilégier ceux qui avaient peu de moyens, distribuant souvent leurs invendus pour les nourrir, sans rien demander, car telle est leur mission morale. Ils n'ont cependant pas été épargnés par les impayés, l'effondrement des ventes et l'impossibilité de stocker une production à très courte durée de vie, quand les charges, elles, sans cesse demeurent. Cette filière a besoin de 1,2 milliard d'euros, de toute urgence, au titre du plan de relance. Elle n'a quasiment rien touché, contrairement à d'autres secteurs, hormis une aide européenne pour la filière viticole. Les effets du confinement sont ignorés dans ce projet de loi de finances pour 2021, alors que la filière a payé au prix fort l'arrêt des commandes liées à la restauration hors foyer.

collectés 143 millions d'euros en 2019. L'objectif, pour 2021, est de 126 millions d'euros. Son avenir est-il donc à la baisse ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer ? Vendredi 27 novembre dernier, les sénateurs de toutes les travées

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le secteur agricole traverse depuis de nombreuses années de profondes difficultés, qui se sont d'ailleurs accrues, pour certaines filières, avec la crise sanitaire : sécheresses et aléas climatiques répétés, répétés, conflits commerciaux, mais également nouvelles charges et contraintes imposées aux agriculteurs. La profession agricole est aujourd'hui habitée par le doute par l'incertitude, alimentés par les injonctions contradictoires de nos politiques publiques et des attentes sociétales. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête de ce ministère, vous portez une voix claire et déterminée de soutien à l'agriculture et à la forêt. nos agriculteurs ont besoin d'être soutenus par l'État, mais ils ont surtout besoin d'une politique et d'une stratégie clairement définies pour le long terme

Ce budget comporte de réelles avancées qu'il convient de souligner. Parmi les plus importantes, je veux tout d'abord saluer la reconduction du dispositif TO-DE, précieux pour les agriculteurs et véritable levier de compétitivité face à la concurrence internationale et européenne. Il est reconduit jusqu'en 2022, alors que sa suppression était prévue fin 2020. À quand sa pérennisation ? Ce budget prévoit aussi le maintien des crédits des chambres d'agriculture et l'abandon du projet de baisse de 45 millions d'euros envisagé l'année dernière par le Gouvernement. C'est une excellente nouvelle, monsieur le ministre. Certes, la revalorisation de la réserve pour aléas, de 175 millions à 190 millions d'euros,

Une fois de plus, selon nous, ce budget est loin d'être suffisamment ambitieux au regard des défis auxquels l'agriculture est confrontée aujourd'hui. La crise du covid-19 nous l'a rappelé : les enjeux de souveraineté alimentaire se font de plus en plus pressants et l'urgence écologique est toujours plus prégnante. Il nous reste très peu de temps pour réagir face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Les moyens proposés sont hélas, à cet

il finance notamment l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), qui réclame à juste titre des moyens à la hauteur de la croissance de cette forme d'agriculture. Je sais, monsieur le ministre,

l'ensemble reste décevant. Les axes du plan de relance qui concernent la territorialisation de l'alimentation et la transition écologique bénéficient d'enveloppes réduites par rapport aux besoins des territoires et par rapport au coeur du plan de relance,

qui contribuent à la fuite en avant du modèle industriel. En effet, les crédits engagés doivent notamment permettre de financer du matériel d'épandage plus précis pour optimiser l'utilisation des intrants. Plutôt que de miser sur des changements de pratiques agronomiques sur des approches territoriales, on finance du matériel. Il y a là surtout un soutien au secteur de l'équipement, au risque d'augmenter l'endettement des fermes et de pérenniser l'usage des pesticides. Cela ne nous convient pas

L'agriculture biologique est la plus performante du point de vue environnemental et économique, comme le rappelle France Stratégie dans son rapport sur les performances de l'agroécologie. La Commission européenne a fixé un objectif de 25 % de surfaces agricoles biologiques pour 2030. Il va falloir mettre le paquet pour y arriver ! Nous sommes d'autant plus méfiants sur la question du soutien à l'agriculture biologique que le Gouvernement a fait le choix d'accorder un financement considérable,

En effet, alors que l'agribashing prospérait assez facilement dans les esprits dans les années 2018-2019, cette crise a rendu à nos agriculteurs toute l'importance qu'ils méritent

font partie de ceux qui ont continué le travail tout au long du confinement afin de nourrir les Français, en général avec fierté et responsabilité. Tous les jours, ou presque, nous le voyons notamment sur les réseaux sociaux, les Français prennent de plus en plus de plaisir à bien s'alimenter, à rechercher le meilleur. Cette appétence pour la bonne cuisine et pour les produits frais et locaux a permis à notre pays de mieux vivre ces moments d'angoisse et d'incertitude. La recherche de la qualité de notre alimentation passe par une exigence citoyenne envers nos produits,

Exigence environnementale, développement des circuits courts, lutte pour le bien-être animal : nul ne pouvait imaginer, il y a encore quelques années, que l'alimentation deviendrait un sujet de société, voire un enjeu politique. Ce gouvernement l'a bien compris et le budget qui nous est présenté est à la hauteur de la situation. Il permet de relever les défis qui ont été fixés dès le début du quinquennat, à savoir améliorer les revenus de nos agriculteurs, assurer notre souveraineté économique tout en renforçant notre compétitivité, enclencher un plan Protéines végétales, développer une alimentation saine et durable, relever les défis climatiques qui, d'année en année, menacent nos exploitations. Ajoutons à ce tableau la reconduction du dispositif TO-DE pour 2021 et 2022. Au total, au titre de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », une fois pris en compte les crédits de paiement du plan de relance, le budget du ministère atteint 3,5 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 13,6 % par rapport à l'année précédente.

représentent au total 455 millions d'euros. Dans quelques semaines, plusieurs dispositifs de soutien à l'investissement matériel seront accessibles aux agriculteurs : aide à l'acquisition de matériel plus performant en matière environnementale,

Ce sujet a alimenté les polémiques médiatiques et a contribué au dénigrement de notre agriculture. Ces polémiques étant vécues comme une profonde injustice par certains agriculteurs, il était temps d'y mettre fin. Ce plan de relance en donne tous les moyens. Ne pas évoquer le récent succès des négociations relatives à la nouvelle PAC n'aurait pas grand sens. Premier budget européen, capable d'orienter les modes de culture et les paysages, cette nouvelle politique agricole commune permettra à la France et à nos agriculteurs de bénéficier de 66,2 milliards d'euros pour les sept prochaines années.

La concertation entre les acteurs du monde agricole permettra de s'entendre sur la déclinaison de la PAC à l'échelon national, à savoir le plan stratégique national (PSN). Ce plan permettra de donner des marges de manoeuvre aux États dans la redistribution des aides européennes. Concernant la déclinaison du premier pilier de la PAC dans nos territoires ultramarins, nous nous félicitons que l'accord de principe obtenu vendredi dernier et confirmé hier par les États membres assure le maintien à son niveau actuel de l'enveloppe du Poséi, le programme Outre le volet agricole, la gestion de la forêt est également un immense défi à relever. Quatrième pays européen en termes de superficie forestière, la France a vu son étendue forestière doubler en l'espace de deux siècles, passant de 9 millions d'hectares en 1830 à 17 millions aujourd'hui.

Ces sommes sont notamment fléchées vers l'ONF, un partenaire essentiel pour notre filière bois, composé d'agents et d'experts passionnés par leur métier. Pour autant, nous le savons, l'ONF connaît depuis quelques années des difficultés importantes, en matière financière, mais aussi de gestion de ses ressources humaines et de dialogue social.

notre groupe votera avec beaucoup d'enthousiasme ce budget qui, en alliant modernisation de notre agriculture et transition agroécologique, vient épauler et accompagner nos agriculteurs afin de leur donner toute latitude pour retrouver rendements, ambition et, surtout, beaucoup de fierté pour le travail accompli.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention venant en complément de celle de Jean-Marie Janssens, je concentrerai mes propos sur le volet forestier de ce programme, pour, une fois n'est pas coutume, saluer les efforts du Gouvernement en matière de soutien à la filière. effort est sans précédent depuis la disparition du Fonds forestier national ; il se traduit- cela a été dit -par la mise en place d'un plan de relance de plus de 200 millions d'euros. Puits de carbone essentiel pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), la forêt est dramatiquement fragilisée depuis quelques années

C'est là un enjeu majeur de ce dossier, monsieur le ministre : notre capacité à fournir les plants dans les essences demandées et dans les temps impartis. Vous avez déjà rendu éligibles à ce fonds les travaux d'amélioration et d'entretien des peuplements jusqu'à 2024. C'était essentiel En effet, pour être efficace, ce plan de relance forestière devra s'inscrire dans le temps long de la forêt et accompagner le suivi des jeunes peuplements. Sans perdre de temps, l'ensemble des professionnels se sont d'ores et déjà mobilisés autour de ces objectifs. Pour autant, certaines problématiques demeurent pendantes et pourraient entraver le bon déroulement de ce plan. Je souhaite donc appeler votre attention sur quelques points. Concernant les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce plan, qui vise à adapter durablement la forêt française aux changements climatiques, pourquoi avoir porté l'obligation de mélange d'essences à 10 hectares, alors qu'il est établi que les mélanges, gage de résilience des peuplements, peuvent se faire à partir de 4 hectares ? Pourquoi ne pas avoir intégré des paramètres relatifs à la densité des peuplements, outil non seulement de résilience face aux déficits hydriques, de gestion des plants face aux problèmes de disponibilité déjà évoqués ? Comment assurer la pérennité de ces reboisements sans organiser une véritable stratégie d'équilibre sylvocynégétique ? Monsieur le ministre, votre capacité à diffuser ce dispositif sur tout le territoire dans les délais impartis dépendra essentiellement de la mobilisation des forestiers, en particulier des agents de l'ONF et du Centre national de la propriété forestière (CNPF) présents sur le terrain. L'Assemblée nationale a déjà réajusté les crédits de l'ONF, permettant le maintien de 95 équivalents temps plein. Dans le même sens, nous vous proposerons un amendement visant à préserver les emplois du Centre national de la propriété forestière. Ses 341 agents interviennent auprès des 3,5 millions de propriétaires forestiers, sur près de 12 millions d'hectares de forêts privées, soit les trois quarts de la forêt française. Pour tous les propriétaires qui ne sont pas adhérents de coopératives, les agents du CNPF sont en effet le principal vecteur de conseils et d'appui au montage des dossiers. Sans leur accompagnement, en l'état actuel des critères d'éligibilité, monsieur le ministre, des milliers de petits propriétaires ne pourront pas avoir accès à votre plan de relance. J'espère donc que vous serez sensible au maintien de ces postes.

L'avenir de l'ONF n'est toujours pas défini ; son déficit grandit et son partenariat avec les communes forestières, le contrat d'objectifs et de performance qui associait les communes, l'ONF et l'État, est aujourd'hui remis en cause, traduisant l'affaiblissement, voire la disparition, d'une stratégie commune de gestion des forêts publiques. L'enjeu, vous le savez, est de taille : il est de mieux faire travailler forestiers publics et privés sur les massifs, au plus près des attentes des populations, pour mieux y répondre. Ce sont là autant de questions qui devront être abordées rapidement pour que votre plan de relance prenne tout son sens et dessine un véritable avenir partagé pour les forêts françaises. Sous réserve de l'adoption d'un certain nombre d'amendements, le groupe Union Centriste optera majoritairement pour un vote favorable sur les crédits

La question est donc de savoir comment et à quoi ces moyens vont être utilisés pour répondre aux enjeux et aux difficultés auxquels l'agriculture française est confrontée. Le budget agricole doit être apprécié à l'aune des questions qui concernent le revenu des agriculteurs et la compétitivité de la « ferme France », l'adaptation aux évolutions climatiques et environnementales et l'évolution du système agricole français, qui s'éloigne toujours davantage du modèle de l'exploitation familiale.

À ce stade, mais vous y reviendrez peut-être, monsieur le ministre, rien n'est prévu en matière d'outils novateurs de gestion des risques. Les besoins en eau, qui devraient être considérés comme une grande cause nationale, sont largement insatisfaits pour faire face à l'avenir immédiat. À ces points problématiques s'ajoute la question du devenir productif de pans entiers du territoire agricole, les terroirs naturellement peu favorisés en termes de qualité agronomique des sols, de conditions pédoclimatiques d'exploitation et, souvent, de topographie. Monsieur Monsieur le ministre, j'ai compris que vous y étiez favorable : il nous faut donner un contenu à la notion de « zones intermédiaires ». Ce qui est en jeu, ce sont les systèmes de polyculture-élevage, qui étaient adaptés à ces terroirs et permettaient aux agriculteurs qui s'y sont succédé des générations durant de vivre correctement. Ce n'est plus le cas et je ne compte plus, chez moi dans le Gers, les exploitants qui disent que tout ou partie de leurs terres ne seront pas reprises. Nos paysages vont se refermer, la nature va reprendre ses droits et nous connaîtrons des problèmes de sécurité publique, comme les incendies ou la prolifération de la faune sauvage.

Il faudra aussi que votre ministère approfondisse l'orientation agroécologique. À cet égard, nous ne comprenons pas le sort qui est fait au Casdar et la volonté manifeste de le faire disparaître par intégration dans le budget général, année après année, alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de financer

Pour terminer, j'appelle votre attention sur la nécessité d'engager un processus législatif concernant la gestion du foncier. Ce qui se joue là, c'est la nature même de notre système agricole. D'année en année, on voit se développer des formes sociétaires, avec des investisseurs, des financiers financiers et une population d'actifs agricoles qui se transforment petit à petit en exécutants. Ce modèle est-il le bon pour le monde paysan ? Est-il gage de vitalité pour les territoires ruraux français ? Je ne le crois pas, et une grande loi foncière serait nécessaire pour traiter cette question d'intérêt national. Au regard des enjeux que je viens d'évoquer, monsieur le ministre, votre action dans les mois à venir nous permettra de porter une appréciation fondée sur votre politique agricole effective.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'aborderai que trois points. Le premier point concerne le coeur de l'action dans nos territoires, à savoir les investissements en agriculture.

nos territoires. On parle de plan de relance, mais on n'a même pas été capable d'accomplir ce qui avait été prévu en termes d'accompagnement des investissements en 2019 et 2020

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année 2020 s'achèvera bientôt, mais la crise sanitaire, économique et sociale est loin d'être terminée. Mes premiers mots seront pour exprimer mon soutien à nos restaurateurs, particulièrement frappés par deux confinements successifs et qui devront attendre la mi-janvier 2021 pour rouvrir leurs portes. Les professionnels de la restauration et de l'alimentation sont directement liés à nos agriculteurs, éleveurs et producteurs, et devront être soutenus « quoi qu'il en coûte ». L'urgence est de prévenir des drames économiques et humains. Comme tous nos concitoyens, nos agriculteurs souffrent de cette situation. Pourtant, au milieu de ce contexte exceptionnel et dramatique, le monde agricole semble avoir mieux résisté que d'autres secteurs économiques. Cela tient notamment à la forte capacité d'adaptation de nos producteurs et au comportement responsable des consommateurs français. Manger bien et local est une réelle priorité pour nos concitoyens et pour notre économie. L'avenir de notre agriculture réside dans cet équilibre entre qualité et proximité. Le projet de loi de finances pour 2021 consacre un budget stable pour notre agriculture. À ce titre, la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » comporte 2,97 milliards d'euros en crédits de paiement, soit 1,1 % de plus qu'en 2020. C'est une nouvelle rassurante pour un secteur essentiel de notre économie et pour l'avenir de nos agriculteurs français. Le programme 149 est d'importance majeure, puisqu'il comprend plus de la moitié des crédits de la mission, soit 1,7 milliard d'euros. Ce programme est particulièrement stratégique. En effet, il a pour objet de structurer et de soutenir les filières, de moderniser et de renouveler les exploitations agricoles et de mettre en place les mesures en faveur de la promotion respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Il est à souligner que le projet de loi de finances pour 2021 alloue une enveloppe de 126 millions d'euros au compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural contre 136 millions d'euros depuis plusieurs exercices. Cette baisse a pour conséquence directe une diminution des budgets des chambres d'agriculture, des instituts techniques agricoles et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Nous refusons cette baisse. Aussi défendrai-je avec plusieurs sénateurs du groupe Union Centriste un amendement visant à stabiliser ces budgets de recherche essentiels pour notre agriculture. Les crédits pour l'année 2021 semblent globalement adaptés aux enjeux de notre agriculture et de ses évolutions. Cependant, il est nécessaire de souligner que l'action menée en faveur de l'agriculture française s'appuie en grande partie sur la politique agricole commune. Or, si la France a obtenu une stabilisation des aides européennes pour notre agriculture, à hauteur de 66,4 milliards d'euros sur la période 2021-2027, des inquiétudes fortes et légitimes planent sur les finalités de cette nouvelle PAC, PAC, notamment en matière de souveraineté alimentaire, de simplification et de concurrence. La politique agricole commune doit servir la qualité, la proximité, la biodiversité, et garantir des revenus justes pour nos agriculteurs. Aussi paraît-il primordial de veiller à ce que la PAC 2021-2027 garde ce cap. Le budget que l'État consacre à l'agriculture française n'aura de sens et d'efficacité que s'il s'appuie sur une politique agricole commune bien conçue et bien articulée avec notre ambition nationale. Le Sénat jouera pleinement son rôle de contrôle et sera particulièrement vigilant et attentif à la mise en oeuvre d'une PAC juste et véritablement bénéfique pour les agriculteurs français.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire n'a pas épargné le monde agricole, qui en sort plus que jamais fragilisé. Inutile de se voiler la face toutefois, l'agriculture française était déjà en souffrance avant même la crise sanitaire. Il en est ainsi de la filière viticole dont je suis issu. Victimes collatérales du conflit sur l'aéronautique entre l'Europe et les États-Unis, ses exportations vers ce pays ont diminué de 35 %. Les restaurants sont fermés, tous les salons sont annulés, les ventes sont à l'arrêt et les pertes financières sont colossales. Ce secteur d'excellence est à genoux. L'aide pour la distillation de crise n'a pas été assez importante, monsieur le ministre. Or, à l'inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises viticoles et agricoles dans leur ensemble n'ont pas eu recours au chômage partiel, étant obligées d'assurer la continuité de la conduite de leur exploitation. Les prêts garantis par l'État souscrits ne pourront être remboursés à court terme. Les mesures de soutien à la filière que vous avez prises n'ont pas atteint correctement leur cible.

Dans ce contexte, le budget pour 2021 était très attendu par la profession, car elle nous demandait des réponses précises, des moyens mobilisables immédiatement. Or les démarches administratives pour l'accès aux aides agricoles sont d'une sombre complexité. Que comptez-vous monsieur le ministre ? Le monde paysan est en grande souffrance. Un agriculteur sur cinq n'a pas de revenu, les jeunes sont endettés jusqu'au cou et les retraités vivent avec des pensions honteuses. Allons-nous continuer à accepter que, chaque jour, un agriculteur se suicide en France ? C'est inadmissible N'avons-nous pas été touchés au coeur par le film, qui a rendu publique la détresse des paysans enfermés dans un système obsolète, que vous avez et que nous avons tous ensemble, ici, la responsabilité de faire évoluer ? Est-il normal que, plutôt que de leur transmettre leurs exploitations, les agriculteurs incitent leurs enfants à changer de métier, laissant place à la spéculation foncière et à la financiarisation de l'agriculture ? La souveraineté alimentaire de la France est mise à mal, la moitié de ce que nous mangeons est importé. La « ferme France » doit évoluer structurellement. Autant vous dire, monsieur le ministre, que nous en sommes encore loin. Répondre à l'urgence est une priorité dans la période actuelle. De ce point de vue, je veux le souligner, votre investissement est très important pour les filières. Le constat est implacable implacable : pandémie, réchauffement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité ... L'heure est grave ! Or, avec les accords de libre-échange, vous engagez nos exploitants sur la voie d'un dumping tarifaire déloyal. Pour compenser la baisse des prix, ils doivent produire toujours plus, dégradant la fertilité des sols et la qualité nutritive des productions. Les ventes de pesticides ont bondi de 25 % l'année dernière et la biodiversité s'effondre. En dix ans, deux tiers des insectes ont déserté les champs, ce qui a un impact à la fois sur la pollinisation

Cela étant, les 1,2 milliard d'euros prévus dans le plan de relance sont une très bonne nouvelle, monsieur le ministre, mais je crains que ce ne soit du ! Pour réussir la transition, il faut du temps. Or, une fois le coup de pouce du plan de relance passé, les efforts risquent de retomber comme un soufflé. Pour conclure, je vous propose de faire de la transition agroécologique un outil de souveraineté alimentaire en investissant prioritairement dans la recherche et l'innovation, afin de repenser nos systèmes agricoles et de protéger la santé des agriculteurs, des consommateurs et de notre planète. La parole

L'une d'entre elles, que nos collègues Françoise Férat, Laurent Duplomb et Jean-Claude Tissot, que je remercie de leur travail, ont à juste titre soulignée dans leur rapport pour avis, est l'inclusion dans le plan de relance d'un volet agricole à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Cette enveloppe répond à l'ambition de réduire le coût des investissements innovants qui permettent d'améliorer le bien-être animal, d'investir dans les abattoirs, de diminuer l'exposition aux aléas climatiques et de réduire l'usage d'intrants. Sur ces 1,2 milliard d'euros, 250 millions d'euros sont consacrés à la modernisation des élevages et des abattoirs. Est-ce suffisant pour sauver des secteurs qui souffrent d'une crise de vocations sans précédent, s'explique à la fois par un manque de rentabilité patent, par des conditions de travail d'une violence inouïe et par un discrédit affligeant, ce que personne ne peut raisonnablement supporter pour moins de 1 000 euros, voire moins de 500 euros Parce qu'elle est plus vulnérable que jamais, je concentrerai mon propos sur la filière viande bovine et ses professionnels, outrageusement caricaturés et présentés comme des criminels par des blasés de tout, sauf d'eux-mêmes. Plus 1,8 % : c'est la hausse de la consommation de viande bovine française depuis le début de l'année par rapport à 2019. C'est bien la preuve que les Français semblent résister à l'utopie ou à la dystopie- à vous de choisir selon votre sensibilité ! -d'une vie sans steak. Pourtant, les cours sont au plus bas. Deux mille : c'est le nombre d'éleveurs bovins, calomniés et harassés, que la France perd chaque année. Si la crise sanitaire secoue bien évidemment la filière, ses difficultés structurelles la mettent au tapis. L'excellent rapport d'information de notre collègue Jean Bizet présenté au mois de juillet dernier détaillait ses problèmes de compétitivité et d'organisation. Son diagnostic était sévère et il prescrivait comme remède l'intervention de la puissance publique. Le Gouvernement propose, quant à lui, 250 millions d'euros pour redresser la barre. Monsieur le ministre, suffiront-ils à diversifier l'industrie de l'abattage et de la transformation ? Suffiront-ils à lutter contre la concentration des centrales d'achat de la grande distribution ? à pallier l'échec prévisible du mirage Égalim, qui n'a pas renversé le rapport de force défavorable aux éleveurs bovins ? Suffiront-ils à mettre au diapason l'offre et la demande de viande de boeuf sur le marché français ? à déployer une véritable stratégie de développement pérenne à l'exportation ? Selon moi, à toutes ces questions, la réponse est « non ministre, que votre ambition n'était pas forcément de résoudre l'ensemble de ces difficultés. Je conçois même qu'elle se bornait à répondre aux cris d'orfraie de quelques militants antispécistes. que, même si nous devions être plus modestes et nous contenter de résoudre l'épineuse question des abattoirs, ces quelques millions d'euros seraient toujours insuffisants. Nous arriverons peut-être à améliorer les conditions de travail épouvantables des employés des abattoirs,

Alors même que ses produits bénéficient d'une réputation de haute qualité, la France doit faire valoir ses atouts sur les marchés extérieurs. Elle doit aussi arrêter de subir un flux croissant d'importations.

le bien-être animal, pour zéro centime de plus sur les cours de vente ces dernières décennies. Monsieur le ministre, c'est à vous et à votre gouvernement qu'il appartient de remédier à ces défaillances économiques, politiques, sociales et sociétales.

monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est à la forêt que je consacrerai mon intervention. La forêt est un bien précieux. Elle représente, derrière les océans, le deuxième plus grand puits de carbone. Elle favorise la biodiversité, protège la ressource en eau, fixe et stocke le carbone. Si elle souffre durement du réchauffement climatique, elle demeure cependant une excellente alliée pour y faire face. Hélas, la vitesse de ce changement s'accélère et favorise le développement de maladies et du parasitisme sur les arbres de nos territoires.

Cette essence est l'une des premières victimes du changement climatique, des épisodes caniculaires et du déficit pluviométrique de ces dernières années. Face à cette menace, il faut une vision à long terme. Il importe d'adapter la gestion forestière, d'évaluer la résistance des espèces et de se tourner vers de nouvelles essences. Toute la forêt française doit faire face à des enjeux similaires. Pour reboiser, il faut des moyens techniques, financiers, humains, à la hauteur des défis qui se présentent. Ces moyens devront être consolidés par des décisions politiques fortes.

Voilà des mesures que nous saluons et soutenons, mais elles sont nécessairement limitées dans le temps, alors que nos forêts exigent de la durée, de la régularité et de la visibilité. Or le budget que nous examinons n'apporte pas assez de souffle face aux besoins de nos territoires forestiers. Par comparaison, nos voisins allemands prévoient 800 millions d'euros entre 2020 et 2023 pour soutenir le reboisement. La politique forestière nécessite des moyens humains et de l'expertise. Or le projet que vous présentiez prévoyait de réduire encore les effectifs de l'ONF. L'Assemblée nationale a rétabli des conditions budgétaires permettant d'annuler cette diminution. Je soutiens Monsieur le ministre, le maintien des effectifs de l'ONF est une nécessité, tout comme le maintien de ceux du Centre national de la propriété forestière, cet établissement public de conseil et d'accompagnement des propriétaires privés, qui exploitent 74 % de la surface forestière. Il me semble essentiel, dans un contexte où la filière bois-forêt est menacée écologiquement et économiquement, de stabiliser les moyens humains dédiés à la forêt.

l'attractivité, la simplicité et l'efficacité du dispositif. Je pense, en particulier, à l'une de ses composantes, le « Defi acquisition », qui doit être assoupli dans ses modalités pour assurer un meilleur regroupement des petites parcelles et faciliter leur exploitation. J'en appelle avec insistance à la pérennisation d'un outil dédié au reboisement, doté de financements à la hauteur des besoins, pour répondre aux enjeux écologiques et développer la filière industrielle du bois.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la forêt représente 31 % de la superficie du territoire. Elle est un atout considérable pour notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la réussite de la transition écologique et économique. Le Gouvernement se félicite d'un plan de relance dédié de 200 millions d'euros. On pourrait croire cette enveloppe généreuse. J'avoue être, pour ma part, beaucoup moins enthousiaste. D'une part, la réduction du nombre de postes d'agents de l'ONF et du CNPF a été unanimement dénoncée par l'ensemble des acteurs du secteur forêt. Je regrette, bien que nos collègues députés aient pu rétablir les effectifs de l'ONF, que ceux du CNPF soient toujours rabotés dans le texte qui nous est présenté, alors même que cet établissement gère, je le rappelle, plus de 70 % de la forêt française.

je sais que la forêt a été sous-dotée- ô combien ! -ces dernières décennies et que le retard à rattraper en termes d'investissement est considérable. Quand je lis, en outre, que nos collègues allemands ont débloqué 800 millions d'euros en faveur de la forêt, je suis inquiet sur notre capacité à exploiter résolument cet « or vert que sur la forme, monsieur le ministre, faites-nous plaisir et modifiez la nomenclature budgétaire ! La forêt mérite un programme dédié, et non une simple action. toutefois de moi l'idée de voir le verre à moitié vide : 200 millions d'euros d'investissement en plus du budget initial, voilà qui représente un premier bon signal pour amorcer la pompe des investissements, qui représentent des recettes pour les communes, des emplois pour nos concitoyens et de l'espoir pour les générations futures. des recettes pour nos communes, car de plus en plus de localités rurales se lancent véritablement dans l'économie forestière. La culture de bois d'oeuvre est un investissement stratégique de long terme, dont les retombées économiques constituent des recettes essentielles pour le fonctionnement des petites communes rurales. des emplois pour nos concitoyens, parce que l'économie sylvicole n'est pas délocalisable. L'économie forestière est une réelle perspective de revitalisation de nos territoires ruraux.

de l'espoir pour les générations futures, car la forêt est le principal levier d'action pour lutter contre le changement climatique. En région Sud par exemple, ce sont 35 % des émissions de CO2 sur le territoire qui sont captées par la forêt et nous visons 50 % d'ici à 2030. L'Accord de Paris nous engage à la neutralité carbone en 2050. La forêt et ses dérivés sont, de loin, notre principal atout pour atteindre cet objectif. Vous le voyez, monsieur le ministre, les attentes sont grandes, les possibilités infinies et votre responsabilité est importante. La parole est à M. le ministre.

Quel gouvernement, y compris du bord politique que vous représentez, monsieur le rapporteur spécial, a consacré 135 millions d'euros pour moderniser les agroéquipements, avec des taux de subvention de 40 % à 60 %- c'est de « l'argent de subvention

L'évaluation des pertes subies par les producteurs de vins et spiritueux mériterait d'être précisée par le Gouvernement, de même que la façon dont l'État a pu les couvrir. J'en profite pour

S'il s'agit d'une première étape importante, cet investissement ne suffira pas pour tirer la commande publique vers le haut et instaurer une boucle vertueuse, car le budget global nécessaire pour la conversion de la restauration collective s'élève à 330 millions d'euros.

Cet amendement traduit la position des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sur la question de la réautorisation des néonicotinoïdes pour la filière de la betterave sucrière. Au mois d'octobre dernier, le Parlement a examiné le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Ce texte vise à réautoriser les néonicotinoïdes jusqu'en 2023 pour cette filière, afin de lutter contre une infestation massive de pucerons vecteurs de la jaunisse. Les sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains se sont opposés massivement à ce projet de loi, qui constitue une régression environnementale majeure. Ils considèrent que le Gouvernement a fait le choix de la facilité en réautorisant un pesticide dangereux pour l'environnement et pour la biodiversité. D'autres réponses auraient pu être apportées à la filière. Comme vous Comme vous l'évoquiez vous-même à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, le 28 juillet 2020, lors des questions d'actualité au Gouvernement, il existait deux solutions : réautoriser les néonicotinoïdes ou mettre en place un soutien financier massif pour la filière afin de compenser les pertes et prévoir la transition. Les parlementaires socialistes plaidaient pour le second choix. Au mois d'octobre dernier, ils ont proposé de mettre en place un plan spécifique mettre en place un plan spécifique visant à sortir la filière de la crise et reposant sur trois piliers : l'innovation commerciale, l'innovation économique et sociale et l'innovation agroécologique. Cette proposition a été rejetée le 30 octobre dernier et un accord a été trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi. Considérant que ce projet de loi ne respectait pas plusieurs dispositions de la Constitution, nous avons déposé, avec plusieurs autres groupes de gauche, un recours devant le Conseil Constitutionnel. Dans l'attente de cette décision

le Gouvernement a souhaité mettre en place des réunions entre citoyens et parlementaires. Si les députés y participent,

vise à accorder une prime à l'investissement permettant aux établissements de s'équiper en matériel, de former leur personnel et de mener des campagnes de sensibilisation, afin d'atteindre les objectifs de la loi

de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d'ici à 2022. Il faut vraiment y mettre les moyens. La restauration collective doit aussi être un levier pour relocaliser notre alimentation.

on continue de trouver des produits importés et de mauvaise qualité dans la restauration collective publique. Nous pourrions pourtant trouver des débouchés rémunérateurs pour nos agriculteurs, avec des produits locaux et de qualité. Il faut engager des moyens pour enclencher une véritable boucle vertueuse. Une fois la transition vers le bio et le local réalisée, le repas ne coûtera pas plus cher. Ces moyens sont de véritables investissements pour l'avenir, dans l'intérêt de nos agriculteurs et éleveurs. à augmenter les financements prévus par le plan de relance de 50 millions d'euros, pour encourager les collectivités à développer une alimentation saine, durable, de qualité et locale dans la restauration collective.

soit toujours de mise, à tous les échelons, pour qu'aucun acquis ne soit perdu dans cette trajectoire vertueuse vers l'autonomie alimentaire et vers la meilleure rémunération des producteurs, sur laquelle nous nous sommes embarqués avec foi et détermination.

De plus, les retards d'application de la promesse du Président de la République, qui s'ajoutent à la crise sanitaire que nous traversons encore, ont renforcé un peu plus la grande précarité de nos agriculteurs. C'est pourquoi, en addition aux 3 millions d'euros qui semblent avoir été ajoutés aux fonds du CIOM, il est nécessaire de soutenir les exploitants agricoles bénéficiaires en augmentant les crédits de 5 millions d'euros supplémentaires, afin d'accompagner au mieux la relance du secteur agricole dans nos régions.

qui estime, dans son rapport, que les « forêts étant indispensables pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour la sauvegarde de notre biodiversité, son entretien et sa surveillance sont primordiaux. Il est donc de ce fait impératif de pérenniser l'existence de l'Office national des forêts

pleinement son rôle face aux défis auxquels sont confrontés nos espaces forestiers, qui sont aujourd'hui mis en péril par le réchauffement climatique et qui font l'objet de fortes attentes sociétales. De plus,

Rien qu'en 2019, ses effectifs ont été amputés de 400 postes, soit d'un emploi sur vingt. Hier encore, dans un article de, on apprenait l'existence d'un projet de filialisation de filialisation des missions d'intérêt général de l'ONF et d'externalisation de leurs travaux forestiers, ce qui conduirait à la suppression de plus de 600 emplois et à la fragilisation supplémentaire de la protection

341 agents permanents pour intervenir sur les trois quarts de la forêt du territoire métropolitain, soit 12 millions d'hectares, et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros. En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement vise également à minorer de 210 000 euros l'action 4, Moyens communs, du programme 215, « Conduite et pilotage des

de maintenir les moyens des deux grands gestionnaires de l'espace forestier : l'ONF, pour la forêt publique, et le CNPF, pour la forêt privée. Les moyens de l'ONF ont été

que du reboisement et du repeuplement de leur parcelle.

l'objectif d'amélioration de la qualité des repas en restauration collective. Le soutien aux producteurs bio est très inférieur à celui qui est demandé. Toutefois,

La conception du Président de la République à ce sujet est très claire : l'Union européenne doit reconnaître la richesse des territoires ultramarins. C'est pour cette raison que le Président de la République s'est beaucoup mobilisé et que nous avons obtenu gain de cause.

pour restaurer la biodiversité du territoire et, enfin, pour relocaliser la production de bois. La forêt française est menacée par le réchauffement climatique, notamment les sécheresses, qui ont entraîné des dépérissements importants. Elle est également frappée par des fléaux sanitaires, liés notamment aux scolytes. Face à ces défis, les montants actuellement prévus par le projet de loi de finances ne sont pas suffisants. Des pratiques de diversification, de recherche et d'expérimentation sur l'évolution de la forêt, des itinéraires techniques alternatifs, le renouvellement par régénération naturelle doivent être soutenus pour permettre le développement d'une forêt résiliente, espace de biodiversité et de production

une tige entourée d'une protection contre les cervidés au milieu de la forêt, c'est que ce n'est pas complètement le produit d'une régénération naturelle ... On peut

Je vous remercie,

n'est plus utilisé.

de développement durable.

monsieur le ministre

Comme je l'ai dit, l'eau doit être une grande cause nationale. Je sais que le Gouvernement y travaille. J'ai apprécié d'entendre M. le ministre exprimer sa résolution politique en la matière. Je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur un sous-sujet

Monsieur le sénateur, vous connaissez ma position sur la question de l'eau : la base de la base, c'est l'eau. Souvent, on se perd dans d'autres débats, faute de courage politique pour affronter le vrai débat de fond, qui est la question de l'eau.

qui subventionne, qui finance, qui aide et qui se montre objective, que de celle de Loire-Bretagne qui fait exactement le contraire. L'argent du contribuable, qui sert aux deux agences, n'est pas utilisé de la même façon. C'est inacceptable dans notre pays.

: La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement vise à créer un fonds spécifique d'aide et d'accompagnement pour aider les agriculteurs à cesser d'utiliser des produits classés cancérogènes probables pour l'homme. Les sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains déposent cet amendement depuis plusieurs années

Ces renoncements ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux actuels et ne permettent pas à nos agriculteurs de prendre clairement le virage de l'agroécologie. Le Gouvernement a certes promis deux enveloppes de 7 millions d'euros pour la recherche d'alternatives au glyphosate et aux néonicotinoïdes,

pérenne afin de cesser au plus vite l'utilisation de pesticides classés cancérogènes probables pour l'homme. Doté dans un premier temps de 10 millions d'euros, ce fonds devra être réévalué en fonction des besoins réels du monde agricole. Quel est l'avis de la commission ? l'avis de la commission ? Cet amendement vise à ouvrir 10 millions d'euros pour accompagner la sortie de l'usage de produits phytosanitaires classés cancérogènes

Le même constat a été établi dans notre assemblée par le rapporteur spécial pour le programme 206, qui souligne « la nécessité d'une réflexion sur les moyens de l'Anses et leur adéquation aux missions de celle-ci, réflexion qui doit aussi considérer les variations du produit

Dans leur proposition, les citoyens demandent une restauration du financement national de l'aide au maintien en agriculture biologique. Je rappelle que, en septembre 2017, le Gouvernement, par la voix du ministre Stéphane

Aujourd'hui, là où les régions n'ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n'ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise le développement de la filière, notamment en élevage. De plus, la nouvelle PAC ne commencera qu'en 2023. Sans soutien national, les exploitations bio

affirme, je le répète, l'efficacité de l'agriculture biologique, définie comme la plus performante du double point de vue économique et environnemental. En 2017, l'aide au maintien représentait 8 à 10 millions d'euros.

monsieur le ministre,

; beaucoup parlé de forêts, et c'est important. Mais votre périmètre, monsieur le ministre, comprend aussi la pêche : il est donc important que nous nous occupions également des problèmes de la pêche,

les plateformes d'initiative locale et d'autres opérateurs susceptibles d'apporter des quasi-fonds propres. Les interventions directes en subventions étant interdites par la réglementation européenne,

Il s'agit d'ouvrir des crédits à hauteur de 5 millions d'euros pour renforcer le contrôle des structures en matière de foncier agricole, afin de favoriser la transmission et le renouvellement des générations.

d'un bien commun dans la durée. Une politique des structures responsable doit privilégier le facteur humain aux dépens du jeu des capitaux et favoriser la diversité au détriment des monopoles : c'est le sens du pacte financier qui, depuis les années 1960, 1960, établit un équilibre entre la propriété et le travail et unit la France à son terroir. Fondée sur la dérive individualiste de la course à l'agrandissement, un relâchement du contrôle, des failles législatives et, depuis 2008, l'arrivée de fonds spéculatifs, une

cela doit nous conduire à nous poser les bonnes questions : si ceux qui nous ont précédés ont trouvé des solutions pour réguler certaines espèces, c'est parce qu'ils subissaient les mêmes dégâts.

nous nous targuons de disposer de la deuxième étendue maritime la plus vaste au monde, nous importons plus de la moitié des produits de la mer que nous consommons. C'est tout de même étonnant

des premier et deuxième piliers de la PAC. Elle est chargée de mettre en place les procédures de gestion et de suivi de paiement des dossiers et de procéder aux contrôles nécessaires. Au vu des difficultés rencontrées depuis des années en matière de versement des aides de PAC et de la mise en oeuvre imminente de la nouvelle PAC, cette diminution ne semble pas opportune et nécessite une explication du Gouvernement. En se fondant sur un montant estimatif de 50 000 euros par ETP, la baisse de 20 ETP pourrait être compensée par 1 million d'euros. Tel est l'objet du présent amendement. Par ailleurs, monsieur le ministre,

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

ne sont pas financés, alors que le Casdar, qui est financé par les agriculteurs, le permettrait. Par exemple, l'Institut technique de l'agriculture biologique est aujourd'hui sous-financé ; une augmentation de son budget le Casdar lui permettrait d'obtenir des fonds complémentaires nécessaires pour accompagner le développement

du programme 775, « Développement et transfert en agriculture », et à majorer de 12,41 millions d'euros l'action n° 01, Recherche appliquée et innovation, du programme 776, « Recherche appliquée et innovation en agriculture

Nous vous avons proposé de nouvelles affectations sur le Casdar ; nous vous avons proposé de reprendre la totalité des financements qui ont été payés par les agriculteurs pour les flécher de façon la plus claire possible